L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2020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 Je rappelle que tous les orateurs, y compris les membres du Gouvernement, s'exprimeront depuis leur place, sans monter à la tribune, et devront respecter les principes de précaution sanitaire

Le Président de la République s'est engagé à déployer tous les moyens nécessaires à la préservation de l'économie de notre pays, du revenu des ménages et des salariés. C'est en effet- l'histoire l'a montré en 2008 -la meilleure façon de faire repartir l'économie

Dès la semaine dernière, nous avons pris des mesures à la fois réglementaires et « d'habitude », afin de permettre aux entreprises qui le souhaitent, en raison de leurs difficultés, de reporter immédiatement leurs échéances fiscales et sociales

pour les collectivités locales -sont à pied d'oeuvre dans des conditions, vous pouvez l'imaginer, très difficiles. Je veux les remercier au nom de la Nation, car eux aussi font marcher l'économie de notre pays. Les mesures de report que nous avons prises représentent une aide directe et immédiate de 35 milliards d'euros, sur les 45 milliards précédemment évoqués : 13 milliards au titre des impôts directs et 22 milliards au titre des cotisations et contributions sociales.

l'article 4 prévoit une garantie exceptionnelle de l'État permettant de soutenir le financement des entreprises à hauteur de 300 milliards d'euros. Ce dispositif temporaire couvrira les prêts accordés du 1 mars au 31 décembre de cette année,

De plus, pour répondre aux inquiétudes des petits entrepreneurs, artisans et commerçants qui subiraient une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des restrictions de circulation et des difficultés liées au coronavirus, le Gouvernement a créé un fonds de solidarité doté de 1 milliard d'euros par mois,

l'initiative du groupe Les Républicains, l'Assemblée nationale a adopté hier un amendement instituant auprès du Premier ministre un comité composé de parlementaires, de représentants des collectivités locales et des entreprises, chargé du suivi et de l'évaluation de la garantie de l'État et du fonds de solidarité des petites entreprises.

cette sage précaution. L'impôt sur le revenu doit être payé par nos compatriotes. Même si, aujourd'hui, c'est l'employeur, le collecteur, qui récupère cet argent, il n'en doit pas moins le reverser dans les caisses de l'État.

Enfin, nous ne laisserons pas tomber les plus petites entreprises, qui sont aujourd'hui les plus durement touchées. Parce que ces entreprises sont les forces vives de la Nation, nous allons mettre en place un fonds de solidarité qui permettra de soutenir les TPE-PME, les indépendants et les micro-entrepreneurs- sous certaines conditions -dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 million d'euros. Des milliers de ces entreprises sont désormais à l'arrêt du fait des arrêtés pris pour préserver la santé des Français et limiter les contacts les contacts sociaux, mais nous n'avons pas le droit de les laisser à leur sort. Le fonds de solidarité aidera également toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires a été diminué de 70

Nous avons décidé d'inclure dans le champ d'application du fonds de solidarité les professions libérales les plus modestes, celles qui pourraient être condamnées par la crise actuelle. Elles seront donc soutenues à hauteur de 1 milliard d'euros par mois, dont 750 millions financés par l'État et 250 millions par les régions.

J'aimerais rappeler à chacun que la solidarité nationale doit jouer à plein régime. C'est pourquoi j'appelle tous les bailleurs privés à faire preuve de solidarité, dès lors qu'ils en ont les moyens. Bien entendu, ces mesures ont un coût pour nos finances publiques. Par conséquent, le déficit public pour 2020 devrait atteindre 3,9 % du PIB, au lieu des 2,2 % prévus initialement. La dette française dépasserait donc 100 % du PIB Les circonstances, exceptionnelles, exigent cette réponse inconditionnelle et puissante. C'est le choix politique que nous faisons. Je salue la décision de la Commission européenne de lever en 2020 les contraintes réglementaires, prévues dans le pacte de stabilité et de croissance (PSC), qui pèsent sur les États membres de la zone euro. La parole

renonce à soutenir les entreprises et les salariés ? Évidemment non ! L'absence de mesures de soutien risquerait d'ailleurs de dégrader durablement les perspectives de croissance de l'économie française. La faiblesse de la croissance va en effet se traduire par une perte de recettes et une augmentation des dépenses sociales. Ainsi, la dégradation de la conjoncture pèse sur le déficit public à hauteur de 1,4 point de PIB. En complément, des mesures de soutien budgétaire à vocation défensive ont été légitimement annoncées par le Gouvernement, afin de permettre aux entreprises et aux travailleurs de surmonter le choc temporaire lié aux mesures de confinement.

appelés à nous revoir ... Au total, la prévision de déficit public s'en trouve d'ores et déjà fortement dégradée, passant de 2,2 % du PIB initialement prévu à 3,9 % à l'issue de l'exercice.

de l'endettement et des mesures de soutien. Il y a néanmoins fort à parier que le scénario gouvernemental sera, de nouveau, substantiellement modifié dans les prochaines semaines. La prévision de croissance constitue naturellement la principale source d'interrogation.

qui pourraient être revues à la hausse en fonction de la durée des mesures de confinement. En outre, il ne peut être exclu que le Gouvernement décide de mettre en oeuvre des mesures de soutien offensives, une fois l'épidémie du

nous en aurons besoin par la suite, mais il s'agit d'un plan de sauvetage. C'est plus tard qu'il faudra aider les entreprises en contribuant à relancer l'économie. Deux mesures sont portées par une nouvelle mission budgétaire intitulée. Les crédits

au niveau mondial, au niveau européen et pour notre pays : l'épidémie de Covid-19 fait des centaines de milliers de malades, des milliers de morts et exige de prendre toutes les dispositions nécessaires pour ralentir et, nous l'espérons, stopper la propagation du virus. Ces mesures fortes et nécessaires ont évidemment une incidence sur notre économie, sur nos perspectives de croissance et sur la situation de nos finances publiques. Par ailleurs, de nouveaux moyens financiers doivent être mobilisés pour soutenir notre système de santé, nos hôpitaux déjà fragiles avant la crise,

soit une dégradation de 2,3 points. Il y a tout juste un mois, alors que notre pays n'était pas encore touché comme aujourd'hui, la dégradation était estimée par le ministre de l'économie et des finances à 0,1 point de PIB. Depuis, la situation a évolué, mais tout peut aussi changer demain si les mesures de confinement se prolongent au-delà d'un mois, si l'environnement économique européen et mondial continue de se dégrader ou si la crise économique se double d'une crise financière. Le Haut Conseil des finances publiques souligne à cet égard un contexte d'incertitude « exceptionnellement élevée ». Il affirme que le scénario du Gouvernement repose sur deux hypothèses fortes, qui ne sont pas acquises : celle d'un confinement limité à un mois et celle d'un retour rapide à la normale de la demande française comme étrangère. Autrement dit, rien ne permet aujourd'hui d'exclure que la chute du PIB ne sera pas plus importante, comme en 2009 lorsque les prévisions n'ont cessé d'être revues à la baisse dans le cadre de plusieurs collectifs budgétaires Bien sûr, on peut se réjouir que la Banque centrale européenne vienne de créer le « programme d'achat urgence pandémique » à hauteur de 750 milliards d'euros, mais les risques demeurent élevés pour les pays européens dont la situation économique et financière n'était déjà pas florissante avant cette crise. Comme je le rappelais dans mon intervention en séance publique le 4 mars dernier, à la fin de l'année 2019, notre dette publique frôlait déjà les 100 % du PIB, contre 60 % pour l'Allemagne, et la France enregistrait le deuxième déficit structurel le plus élevé de la zone euro. Alors que nous avons profité jusqu'à présent d'une charge de la dette allégée grâce aux taux d'intérêt bas, celle-ci risque de fortement remonter. Le déficit public devrait, selon l'estimation du Gouvernement, atteindre 3,9 % du PIB fin 2020 contre une prévision de 2,2 %, soit une hausse de 15 milliards d'euros. Cela résulte des mesures nouvelles de soutien qui s'élèveraient à 11,5 milliards d'euros- dont 8,5 milliards d'euros pour la mise en activité partielle -, mais aussi de la chute des recettes fiscales de 10,7 milliards d'euros, particulièrement celles de l'impôt sur les sociétés et la TVA. Cependant, l'incidence de la crise sur les dépenses budgétaires et les recettes fiscales pourrait être très largement supérieure si la crise perdure. De manière complémentaire, les mesures pour répondre au choc économique pourraient se révéler insuffisantes. Des secteurs économiques souffrent fortement, comme ceux de la restauration, de l'événementiel, des spectacles, de la culture. D'autres, comme une partie du commerce, le transport aérien, le tourisme, risquent de souffrir aussi très fortement, très subitement et très durablement de cette situation. Le fonds de solidarité pour les très petites entreprises en difficulté, cofinancé par les régions, est bienvenu, mais il paraît très sous-dimensionné

J'estime que la crise économique qui s'annonce, avec la baisse de nos recettes fiscales, devrait nous amener à reconsidérer les très importants allégements de fiscalité pour les détenteurs des plus hauts patrimoines. Les revenus en flux seront affectés, en forte baisse. Il sera donc difficile de les surtaxer. Mais les revenus en stock, c'est-à-dire liés à un capital détenu, restent possiblement contributeurs. Certes, les marchés financiers sont en baisse, mais notre nation a plus que jamais besoin de la solidarité de tous et nous devons mobiliser celles et ceux qui sont le plus capables de contribuer aux efforts collectifs, surtout si l'on garde à l'esprit les importants allégements de fiscalité-ISF et prélèvement forfaitaire unique (PFU)-que nos récents travaux parlementaires ont permis de révéler En conclusion, ce collectif budgétaire n'est qu'une première réponse, très immédiate, à la crise. Il sera suivi nécessairement d'autres mesures. La crise que nous vivons aujourd'hui est inédite par sa soudaineté et par son ampleur. Pour qu'elle ne s'aggrave pas davantage, il faudra, au-delà de nos mesures nationales, que l'ensemble des pays européens adoptent des dispositifs forts de soutien à l'activité et fassent preuve de solidarité, notamment à l'égard des pays les plus fragiles, afin de ne pas risquer une déstabilisation de nos économies.

monsieur le ministre, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, depuis plusieurs semaines déjà, la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus s'est doublée d'une crise économique et financière. Ce contexte nous oblige désormais à reconsidérer toutes les hypothèses en fonction desquelles nous avons voté, il y a trois mois seulement, la loi de finances initiale. Depuis les mesures d'urgence prises par le Gouvernement afin de limiter les déplacements de nos concitoyens, et donc de ralentir la circulation du virus, l'économie tourne au ralenti : consommation en forte diminution, stabilisation des investissements, contraction du commerce international La récession est désormais certaine, alors que nous avons bouclé, voilà quelques mois, un budget établi sur la base d'un taux de croissance supérieur à 1 % du PIB. En conséquence, toutes nos prévisions financières doivent être C'est un état de fait. Ce projet de loi de finances rectificative en prend acte. Et la réalité qui y est décrite est malheureusement alarmante : le déficit public, que nous parvenions à peine à maintenir sous la barre des 3 %, bondira en 2020 à 3,9 % du PIB. Cela ne fait aucun doute : les efforts financiers proposés par le Gouvernement sont nécessaires. La France ne peut pas en faire l'économie. Bien sûr, pour d'autres pays, qui ont mené ces dernières années des politiques très ambitieuses et courageuses de réduction des dépenses publiques, ces efforts seront plus accessibles. Mais soyons-en certains : face à l'urgence de la situation, le doute ne nous est pas permis. Nous devons agir rapidement et efficacement. Il faut que l'État prenne les mesures adaptées à l'urgence de la situation, quoi qu'il en coûte. Mon groupe votera ce projet de loi de finances rectificative. Nous espérons que les mesures prévues ne dégraderont pas le déficit structurel et qu'elles soutiendront utilement nos entreprises. Cependant, une fois que nous aurons vaincu le virus, une fois que nous aurons su relancer l'activité de nos entreprises, notre regard sur la résilience économique de notre pays aura changé. Il y aura bien un avant et un après cette pandémie en matière de stratégie économique. J'envisage, pour ma part, deux axes de réflexion structurants. Le premier concerne la relocalisation de certaines activités stratégiques. Nous avons récemment pris conscience de la dépendance à l'international de secteurs de souveraineté. Or cette dépendance a aujourd'hui de lourdes conséquences, tant sur nos comptes publics que sur nos entreprises. Elle obère notre capacité à réagir rapidement en situation de crise. Le second a trait à nos contributions au projet européen. Nous avons également pris conscience, au cours de cette crise, de l'importance d'une action coordonnée à l'échelon européen. Nous aurons besoin de plus d'Europe pour défendre les intérêts de la France, car les crises du XXI siècle, comme celle que nous traversons aujourd'hui, ignoreront les frontières nationales. C'est ensemble, et avec l'unité de toute la Nation, que nous surmonterons cette épreuve.

nous voyons de quoi sont capables les médecins, les infirmiers et les aides-soignants. Au nom de l'ensemble des membres du groupe Union Centriste, je tiens à leur faire part de notre admiration et à leur adresser nos remerciements les plus chaleureux. Nos pensées accompagnent également les policiers et les gendarmes, ainsi que tous ceux qui font fonctionner les services publics et tous ceux qui demeurent actifs dans notre économie, en particulier dans les filières d'approvisionnement. C'est dire que le Sénat dans son ensemble et le groupe Union Centriste en particulier abordent ce PLFR avec esprit de responsabilité. Nous souhaitons aboutir vite à une vision commune avec le Gouvernement et l'Assemblée nationale, et nous savons déjà que ce projet de loi de finances rectificative sera inévitablement suivi d'autres. Nous saluons la réactivité du Gouvernement et l'ampleur financière des mesures déployées, que justifient la gravité et l'urgence de la situation. Afin d'amortir au mieux le choc économique et financier créé par l'épidémie de coronavirus, choc dont on peine à mesurer toute l'étendue, l'État doit déployer sans tarder l'artillerie lourde, faite d'une palette diversifiée de mesures qui vise à ne laisser aucune entreprise ni aucun ni aucun particulier au bord du chemin ... Le défi est gigantesque par son ampleur. Nous devons parvenir à ne pas gripper les filières d'approvisionnement, à sauvegarder les compétences et les savoir-faire- d'où le chômage partiel -, à maintenir la capacité productive et le tissu économique, mais nous devons aussi parallèlement veiller à la solidité financière de l'État. Cette double exigence- faire face aux effets de la crise sanitaire et en même temps préserver la solidité financière de l'État -constitue un immense défi. Il ne faut pas qu'une crise financière propre à l'État aggrave encore les difficultés du pays. De ce point de vue, le niveau des taux d'intérêt et la capacité à financer notre dette lors de chaque émission doivent rester des marqueurs. Il faut d'abord faire face aux difficultés nées de la crise sanitaire que nous traversons. Cela a été dit, les 45 milliards d'euros du plan de sauvetage à effet immédiat permettront de financer tout à la fois le report des charges fiscales et sociales des entreprises, le renforcement du dispositif de chômage partiel, le paiement d'indemnités journalières, ainsi que le fonds d'indemnisation pour les indépendants et les commerçants. De la même manière, la garantie des prêts bancaires accordés aux entreprises à hauteur de 300 milliards d'euros doit permettre aux banques d'octroyer facilement des prêts aux entreprises qui se trouveront ou se trouveraient déjà en difficulté. La conséquence de ces mesures et de celles qui immanquablement suivront sera une dégradation lourde, mais inévitable, de nos finances publiques. Cette dégradation est sans doute sous-évaluée à ce stade, mais comment faire autrement ? Mécaniquement, les nouvelles prévisions budgétaires pour 2020 se dégradent. Le déficit budgétaire, qui se détériorerait de 15,4 milliards d'euros, est ainsi revu à 108,5 milliards d'euros pour la fin de l'année. C'est là, monsieur le ministre, une estimation qui nous paraît quelque peu optimiste Le niveau du déficit serait alors sensiblement équivalent à celui qu'avait déjà retenu le ministère de l'économie et des finances à la fin de l'année 2018, dans le sillage de l'annonce des mesures destinées à répondre à la crise des « gilets jaunes ». Or le séisme nous semble cette fois-ci relever d'une intensité et d'une magnitude autrement plus importantes La baisse à hauteur de 10,7 milliards d'euros des recettes fiscales, supportée aux deux tiers par l'impôt sur les sociétés, est parfaitement intelligible. En revanche, peut-on assurer raisonnablement, comme le suggère l'exposé des motifs du présent PLFR, que la hausse des dépenses du budget général de l'État sera à peine supérieure à 6 milliards d'euros ? Pour indispensables qu'ils soient, les crédits immédiatement débloqués pour freiner la propagation du coronavirus appelleront de nombreuses autres dépenses à la chaîne, pour l'heure peu prises en compte D'après certains conjoncturistes, et sur la base d'un scénario conventionnel calqué sur le scénario de sortie de crise postérieur à 2008, notre ratio de déficit public pourrait durablement franchir la barre des 4 voire celle des 5 %, celui de l'endettement dépassant même la barre des 115 % du PIB à l'horizon de 2024. Et encore un tel scénario repose sur une stabilisation du déficit structurel à son niveau de 2019 Si maintenant nous essayons de nous projeter dans cet avenir incertain, il paraît inévitable qu'un plan de relance succédera, lorsque le virus sera moins actif, à ce plan de sauvetage. Nous pouvons nous féliciter que les mécanismes européens permettent de dépasser l'horizon des 3 %. Sans doute y a-t-il dans la définition de politiques communes à l'échelle européenne des voies de solution pour l'avenir. Les initiatives prises vont dans le bon sens. Il faudra tirer le moment venu toutes les leçons de cette crise terrible. Il faudra bien sûr financer plus et mieux le régalien, au premier rang duquel le système

Nous sommes nombreux à avoir lancé l'alerte et à avoir souligné qu'en cas de crise subite les marges de manoeuvre financières manqueraient. Nous y sommes ! La crise du coronavirus doit nous inviter à revoir nos priorités et à engager enfin structurellement la réforme de notre appareil d'État, maintes fois différée La lucidité doit être le premier de nos courages. Tôt ou tard, et mieux vaudrait tôt que tard, il faudra avoir la force d'admettre que notre capacité à surmonter les défis n'est pas corrélée à celle de dépenser toujours plus, mais à celle de dépenser mieux. Dans l'immédiat, le groupe Union Centriste se félicite de la radicalité des mesures prises par le Président de la République et le Premier ministre. Il faut un soutien radical de l'État pour sortir le pays d'une situation radicalement bloquée. C'est évidemment dans cet esprit que nous voterons pour le présent projet de loi de finances rectificative,

cela témoigne de l'extrême fragilité de nos sociétés, voire de notre civilisation. Face à cette crise sanitaire inédite, par son mode de diffusion plus, peut-être, que par sa gravité, le Gouvernement, comme dans de nombreux pays touchés, se trouve dans l'obligation de réagir dans l'urgence. À cet égard, je tiens à saluer la réactivité dont il a fait preuve ces derniers jours en prenant des mesures d'application immédiate de prise en charge du chômage partiel et de report du paiement des charges sociales et fiscales au 15 mars. L'économie française va être confrontée à un double choc : un choc de la demande, sans doute suivi d'un choc de l'offre. Elle doit faire face à un niveau d'incertitude élevé quant à la durée et à la persistance des effets de ces

Bien sûr, les dépenses budgétaires vont augmenter et les recettes diminuer, le déficit public et l'endettement vont s'accroître. Ce scénario est inévitable pour l'année 2020. Les chiffres qui nous ont été communiqués aujourd'hui ne peuvent avoir qu'un caractère provisoire et me semblent, d'ailleurs, relever d'une approche un peu, peut-être trop, optimiste. Peu importe : nous serons amenés à les revoir de manière mieux documentée dans les semaines et les mois à venir. L'important, ce sont les mesures prises pour faire face à une crise économique naissante qui risque de se répandre à la même vitesse que le coronavirus lui-même. Notre appareil économique est en effet menacé d'affaiblissement, voire, dans certains secteurs d'activité, de destruction. Les mesures annoncées en faveur des entreprises et des salariés vont dans la bonne direction, mais leur efficacité dépendra de la déclinaison qui en sera faite, secteur d'activité par secteur d'activité, entreprise par entreprise. Elles doivent à la fois traiter le présent et préparer l'avenir, être souples et adaptées dans leur mise en oeuvre, tout en préservant des conditions équitables de concurrence. Les facilités accordées aux entreprises ne doivent pas consister en un décalage de quelques mois du paiement des charges sociales et fiscales

Le dispositif exceptionnel de garantie permettant de soutenir le financement bancaire des entreprises à hauteur de 300 milliards d'euros est un excellent outil, dès lors que sa mise en oeuvre est contrôlée par un opérateur public, en l'occurrence

détournent l'esprit de cette mesure pour garantir des prêts ordinaires dans ce dispositif. Je fais plus confiance à Bpifrance qu'à l'ensemble du secteur bancaire

Il est préférable de prévoir une période blanche de remboursement en capital et un allongement équivalent de la durée du remboursement du prêt. Enfin, je veux attirer votre attention sur la nécessité de préserver une équité de concurrence entre les entreprises, en particulier dans le secteur de la distribution.

établir des règles. Telles sont les quelques réflexions ou contributions que je voulais vous livrer, au-delà de l'aspect purement budgétaire, qui est essentiel, mais dont l'urgence est peut-être moins grande que la mise en oeuvre de mesures de soutien destinées à sauver notre économie. Même si nous allons examiner quelques amendements, lesquels, s'ils peuvent présenter un intérêt, ne sont peut-être que des amendements d'appel, je souhaite que ce texte puisse être voté conforme : cela constituerait le meilleur encouragement que nous pourrions adresser à nos entreprises et à leurs salariés. La

pour sauver des vies et faire reculer le nombre de contaminations. Je salue nos forces de police ainsi que les pompiers, qui ne comptent pas non plus leurs heures, comme les agents de vos ministères et ceux du Sénat, qui nous permettent de fonctionner aujourd'hui.

Il est donc primordial de réagir puissamment sur le volet économique et budgétaire. Ce projet de loi de finances rectificative est un bouclier fiscal et budgétaire pour répondre au choc économique qui s'amplifie avec la crise sanitaire en cours. Il est également en lien avec les décisions prises par la Banque centrale européenne pour sauver la zone euro. Il s'agit non plus aujourd'hui de ferrailler sur les ratios budgétaires ou de polémiquer sur les crédits, mais d'apporter la réponse adéquate pour protéger nos compatriotes et pour sauver nos entreprises. Nous savons que ce budget est une première réponse et que d'autres textes financiers pourraient suivre, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Cette première réponse est massive

Ces circonstances exceptionnelles justifient l'écart avec les trajectoires budgétaires habituelles, comme l'a reconnu le Haut Conseil des finances publiques. Il ne faut pas agiter le boulier quand la Nation a besoin d'un bouclier.

il faudra profondément revoir nos modalités d'action. Cela vaut, bien sûr, pour notre système de soins, notre solidarité du quotidien, les avancées de notre recherche, notre autonomie alimentaire et notre souveraineté industrielle. Bref, il s'agit non pas de faire de la science-fiction, mais de refonder les politiques publiques. Je ne prendrai qu'un seul exemple : c'est l'occasion d'approfondir la transition numérique pour être davantage prêt la prochaine fois. Télétravail, télémédecine, cours en ligne pour nos enfants, visioconférence, y compris au Parlement : nous allons devoir apprendre à fonctionner de manière différente. Il faudra également développer le scrutin électronique dans notre pays. Soutenir nos entreprises, de toutes tailles, dans cet épisode de turbulences, est indispensable. C'est une dépense exceptionnelle, mais, à long terme, rien ne sera plus comme avant cette guerre. Je le pense profondément. Nous devons sortir transformés de cette crise : les règles budgétaires devront aussi être réévaluées à cette aune, en distinguant davantage ce qui relève du fonctionnement et de l'investissement et en nous attachant, surtout, à la qualité des dépenses publiques plus qu'aux ratios quantitatifs exprimés en pourcentages. Dans un monde incertain, instable, imprévisible, les vieilles habitudes n'ont plus cours ; il faut investir pour préparer les crises et définir les nouvelles règles du jeu qui vont avec les nouveaux risques. Il faut redonner de l'espoir à nos enfants et refaire Nation. Je termine en paraphrasant un vers de Guillaume Apollinaire, qui a été emporté par une autre pandémie

Mon groupe part de ce point de vue : nous devons examiner les propositions qui nous seront faites en termes économiques et financiers au regard de l'état d'urgence sanitaire

du surendettement du secteur privé. N'avons-nous plus de mémoire ? Il n'y a plus de rachat d'actions, plus de fusions-acquisitions, plus d'opérations spéculatives ? Il faut qu'on parle franco aux Françaises et aux Français,

face à la crise sanitaire sans précédent que vit notre pays, avec pour corollaire un impact potentiellement très grave sur nos entreprises et notre pouvoir d'achat, les mesures d'urgence décidées par le Gouvernement, visant à sauvegarder notre économie, nécessitent de voter ce collectif budgétaire, pour en garantir le financement, à travers, notamment, l'ouverture des crédits nécessaires. Autant le dire tout de suite, le groupe Les Républicains votera bien évidemment ce texte. Nous regrettons que le Gouvernement n'ait pas fait ces trois dernières années les efforts nécessaires pour dégager des marges de manoeuvre budgétaires, contrairement à la plupart de nos voisins européens, mais mon collègue Philippe Dominati reviendra sur ce point au cours de son intervention. estimons pourtant que, à ce stade, le Gouvernement est globalement à la hauteur dans les réponses qu'il apporte à la crise. Par expérience de la crise de 2008, nous savons qu'il faut répondre vite et fort. Toutefois, ce collectif budgétaire tend seulement à sauvegarder, dans l'urgence, notre économie. Monsieur le ministre, confirmez-vous qu'il sera suivi d'un prochain collectif d'ici à l'été, visant cette fois-ci à relancer l'économie ? Les nouvelles prévisions contenues dans le texte que nous examinons aujourd'hui, que nous jugeons plutôt optimistes, seront alors très certainement de nouveau révisées, en fonction de l'évolution de la situation. Pour le moment, les prévisions pour 2019 et le déficit structurel pour 2020 restent inchangés par rapport à la loi de finances pour 2020. Le déficit provisoire de l'année 2019 sera publié par l'Insee à la fin du mois de mars. En revanche, le très fort ralentissement économique lié au double choc de l'offre et de la demande, consécutif aux mesures de lutte contre l'épidémie du coronavirus, constitue un effet de ciseaux inédit et redoutable, qui va entraîner une chute du PIB, dont l'évolution est reprogrammée de +1,3 dans la loi de finances pour 2020 à-1 %, soit une perte de 2,3 points ! Lors de la dernière crise économique et financière, le PIB avait chuté de 2,6 points de +0,3 % en 2008 à-2,9 % en 2009. Ce ralentissement de l'économie va entraîner une chute des recettes fiscales en 2020, de 10,7 milliards d'euros : une baisse, notamment, de 6,6 milliards d'euros de l'impôt sur les sociétés, de 1,4 milliard d'euros de l'impôt sur le revenu et de 2,2 milliards d'euros de la TVA. Je rappelle que, dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale, qui entrera en vigueur en 2021, mon groupe avait alerté le Gouvernement sur le risque de faire reposer l'essentiel des recettes fiscales des départements sur la TVA, très sensible à la conjoncture, et alors même que les conseils départementaux sont en première ligne en matière de dépenses sociales, en cas de retournement conjoncturel. Nous en avons l'illustration Le déficit public va, en conséquence, s'envoler, de 2,2 % prévus par la loi de finances pour 2020 à 3,9 %. Cette prévision est d'ailleurs provisoire et sera probablement révisée à la hausse, car elle repose sur une hypothèse optimiste de sortie de crise et ne tient pas compte des futures mesures de relance. D'ores et déjà, les mesures d'urgence et de sauvegarde vont entraîner une explosion de la dépense publique, qui sera financée par la dette publique, laquelle va dépasser très largement le cap des 100 % du PIB en 2020. Les mesures d'urgence s'élèvent au total à 45 milliards d'euros. Toutefois, près de 35 milliards d'euros prennent la forme d'une avance de trésorerie, puisqu'il s'agit du report pour les entreprises du paiement des charges sociales et des impôts : 12 milliards d'euros pour l'impôt sur les sociétés, 13 milliards d'euros pour les charges sociales dues par les grandes entreprises au 5 avril, 8,5 milliards d'euros pour les charges sociales dues au 15 mars et 1 milliard d'euros pour la taxe sur les salaires. Sur ce point, nous regrettons très fortement que la TVA ne soit pas concernée. Ces 35 milliards ne devraient donc pas, au final, affecter les finances publiques. Demeurent plus de 10 milliards d'euros de dépenses non remboursables, prévues pour les deux prochains mois, dont, notamment, 5,5 milliards d'euros d'indemnisation du chômage partiel, 2 milliards d'euros pour le fonds de solidarité pour les TPE et les indépendants, avec une première participation des régions de 250 millions d'euros, et 2 milliards d'euros de dépenses de santé, soit le paiement des arrêts maladie, d'assurance maladie), l'achat de masques, le versement des indemnités journalières et les mesures de reconnaissance pour le personnel médical. Sur ce point, mon groupe regrette que l'Assemblée nationale n'ait pas adopté un amendement visant la défiscalisation et la désocialisation des heures supplémentaires. Le personnel médical, les forces de l'ordre, les magasiniers, tous les Français qui ne comptent pas leurs heures en ces temps difficiles pour tenter de maintenir le paquebot France à flot et sont parfois épuisés, méritent d'être encouragés. Notre rapporteur général déposera un amendement similaire et nous espérons que le Sénat, dans son ensemble, le votera. Les mesures d'urgence que j'ai détaillées constituent des dépenses : elles sont calculées pour les mois de mars et d'avril, mais s'y ajouteront les futures dépenses du plan de relance économique qui devra être mis en oeuvre après la crise. De surcroît, les reports de paiement d'impôts et charges, qui sont aujourd'hui de simples mesures de trésorerie, pourront se transformer en annulations dans certains cas, comme l'a laissé entendre Bruno Le Maire. Tout cela s'entend sans compter, pour les comptes publics, les dépenses des collectivités territoriales : les communes et les départements pour les aides sociales, ainsi que les régions pour les aides économiques. Le coût de la crise pour les finances publiques devra aussi tenir compte des baisses importantes de recettes fiscales, qui pourraient être aggravées par une élasticité des recettes supérieure à un, comme c'est souvent le cas en période récessive, alors que le Gouvernement prend comme hypothèse optimiste une élasticité de 1. Le Haut Conseil des finances publiques, dans son avis du 17 mars 2020, souligne d'ailleurs que le PLFR repose sur des hypothèses « d'une grande fragilité » : un confinement pendant un mois seulement et une reprise rapide de la demande. Il estime que la dégradation de la situation macroéconomique pourrait être plus importante que ce qui est prévu dans le présent texte. Pour financer les mesures du Gouvernement, la France va notamment lever 5 milliards d'euros de plus d'obligations à moyen et long terme sur les marchés en 2020, portant le montant total des émissions à un nouveau record de 210 milliards d'euros. C'est du jamais vu Par ailleurs, le collectif budgétaire prévoit une mesure de sauvegarde importante, que nous approuvons : une garantie de l'État relative aux prêts consentis par les banques aux entreprises. Assurée du 16 mars 2020 au 31 décembre 2020, elle atteint 300 milliards d'euros. Elle est gérée par Bpifrance, qui garantira donc jusqu'à 90 % des prêts bancaires, alors que le seuil habituel de garantie est de 50 %. Ce dispositif doit permettre de rassurer les banques, afin que ces dernières continuent d'accorder des prêts aux entreprises pendant la crise, pour faire face, notamment, aux conséquences de celle-ci. En cas de difficulté de l'entreprise, la banque prêteuse ne supportera que 10 % du risque. Le montant de la garantie est dimensionné par rapport à l'encours total de crédits aux sociétés non financières, à hauteur de 1 063 milliards d'euros en janvier 2020, dont 240 milliards d'euros de crédits de trésorerie. Notons, en outre, que cette garantie nationale est complétée par 1 000 milliards d'euros de garanties de prêts bancaires dans la zone euro, dont l'Eurogroupe a décidé l'engagement ce 16 mars 2020. Les prêts visés devront répondre à un cahier des charges et ne pourront pas concerner des entreprises en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation. La garantie publique n'est pas actionnable sur les procédures collectives. Ces conditions visent à réduire le risque financier pour l'État de voir une partie des 300 milliards d'euros engagée en cas de défaillances d'entreprises dont il aura garanti les prêts bancaires. Les banques pourront alors en effet y faire appel. Ce panel de mesures constitue indéniablement une première réponse à la crise sans précédent que nous traversons. Comme je l'ai déjà exprimé, mon groupe les votera sans hésitation. Il y va de la sauvegarde de notre économie. La parole

Cela nous paraît nécessaire, car, pour le dire très directement, nous ne sommes absolument pas convaincus que la crise prendra fin dans un mois, compte tenu de l'expérience que nous avons de la récession de 2008-2009. Encore une fois, l'urgence à agir fait que nous ne rajouterons pas de la crise à la crise, ce serait irresponsable. Mais je veux utiliser ce temps de discussion générale pour vous alerter sur les réserves qui sont les nôtres. L'actualisation de vos prévisions macroéconomiques de l'article liminaire sera nécessaire, dont acte. L'avis du Haut Conseil des finances publiques est très explicite, comme l'a rappelé le président Éblé. Il confirme cette inquiétude et l'ampleur des impacts inédits auxquels nous aurons à faire face collectivement. Je mesure les délais contraints de travail qui ont été les vôtres et ceux de votre administration, monsieur le secrétaire d'État, que je veux d'ailleurs saluer, ainsi que les personnels soignants, les fonctionnaires, les salariés du privé qui, partout sur le territoire national, incarnent la continuité de l'État et sont indispensables au fonctionnement de notre vie quotidienne. Le moment venu, il ne faudra pas l'oublier. Votre projet de loi de finances rectificative repose sur un plan de 45 milliards d'euros injectés dans l'économie nationale, déployant des avances de trésorerie indispensables pour la survie de notre économie et l'engagement de nouvelles liquidités.

Je ne doute pas que ces 2 milliards soient bien quelque part ... Je vous invite à faire attention aux effets d'annonce qui ne sont pas pleinement opérationnels ou dont chacun de nos concitoyens ne peut constater la véracité et les effets. J'en viens maintenant à deux articles du projet de loi de finances rectificative dans lesquels on constate tout d'abord la création d'une mission budgétaire- pourquoi pas ? Je ne suis pas convaincu qu'un tel dispositif soit le plus à même de mobiliser l'ensemble des administrations publiques dans le combat que nous devons conduire, mais il aura le mérite d'unifier les canaux de décision,

nous soutiendrons bien évidemment ces mesures, car elles sont nécessaires. Mais il y a plus important en la matière : vous réajustez les prévisions fiscales et, par voie de conséquence, les équilibres de la mission « Remboursements et dégrèvements ». C'est fort logique, même si, là encore, il faudra très vraisemblablement reprendre toutes les estimations encore trop incertaines. Rien sur la mission « Santé », ce qui ne peut que surprendre. Rien non plus, ce qui fausse grandement nos prévisions macroéconomiques selon moi, sur la mission « Engagements financiers de l'État alors que l'on constate une légère remontée des taux, même si la signature de la France est certaine, comme l'a rappelé M. Darmanin à l'instant et comme l'ont prouvé les dernières émissions de jeudi. Le besoin de financement de l'État, à ce stade, s'élève à près de 246 milliards d'euros. d'euros. Aux 45 milliards annoncés, qui ne représentent, il est vrai, qu'environ 8 milliards d'euros de réelles dépenses, il faudra sans doute ajouter le paiement d'intérêts. Je serai bref sur l'article 3 portant sur les comptes spéciaux. Le renoncement à la vente d'Aéroports de Paris, ce qui est une très bonne chose, se traduira par une recette en moins pour l'État et par des dépenses équivalentes, sachant que 2 milliards d'euros étaient affectés au désendettement de l'État. Il serait opportun d'avoir des précisions sur la valeur qui était alors attendue de la cession d'Aéroports de Paris.

que ce vote, motivé par les enjeux d'urgence, ne constitue nullement un blanc-seing au Gouvernement. Il convient que le Parlement soit associé et puisse contrôler le Gouvernement. En ce sens, les propositions du rapporteur général sont intéressantes. Je voudrais conclure mon propos en rappelant que ce texte financier est extrêmement atypique, pour ne pas dire unique, en ce qu'il prévoit- c'est logique -des dépenses sans proposer de recettes. Mais je ne doute pas que cela viendra., dans l'urgence, les réponses à la crise se font par le creusement de la dette. Le pacte de stabilité- c'est une bonne chose -est suspendu. La décision de la BCE est bienvenue. Toutefois, je tiens à rappeler que l'instauration d'une imposition sur le revenu en France, par le biais de la loi Caillaux, date de 1914. Après sept années de débats parlementaires qui n'avaient pas permis de trouver une solution satisfaisante, c'est l'entrée en guerre de la Nation qui a conduit les parlementaires à accepter la mise en oeuvre de tels prélèvements fiscaux. À l'heure actuelle, nous sommes en guerre, comme l'a répété le Président de la République. Dès aujourd'hui, nous devons donc préparer le jour d'après que nous espérons très prochain. Je souhaite, au nom du groupe socialiste et républicain, que notre pays puisse dépasser dans la solidarité cette épreuve.

et, à l'instar de ce que réclame le Medef, de réinjecter ces sommes, au nom de la solidarité nationale, dans le plan de relance économique à venir pour soutenir l'activité et l'emploi dans le prolongement des propos tenus par le président de la commission des

la France connaît actuellement sa plus grave crise sanitaire depuis un siècle. Le coronavirus circule sur notre territoire national. Il constitue une menace dont l'ombre grandit chaque jour. Mais au-delà de la situation sanitaire, laquelle doit demeurer notre priorité absolue et notre seule boussole pour lutter contre le virus, la situation économique et financière s'avère d'ores et déjà très préoccupante. Je pense à toutes nos entreprises, tout particulièrement à nos TPE et PME, qui doivent faire face à des difficultés nouvelles qu'il faut traiter dans l'urgence, comme les annulations en cascade de leurs commandes, les difficultés d'approvisionnement et de financement ou la réorganisation contrainte de leurs ressources humaines. Nous devons maintenant les rassurer et les accompagner avec des outils adaptés, efficaces et réactifs. Le Gouvernement propose des mesures d'urgence, à savoir le renforcement du dispositif de chômage partiel pour l'accompagnement des entreprises dans la gestion de leur force de travail, la garantie apportée par l'État à toutes les entreprises en difficulté demandant un crédit et des reports de charges et d'un certain nombre de modalités fiscales. travers cette crise, nous reprenons conscience de tout ce que l'État peut apporter aux acteurs économiques un filet de sécurité, une garantie collective contre les crises imprévisibles, un soutien pour accompagner les acteurs français dans la tourmente mondiale- je pense notamment à la garantie apportée par l'État grâce à Bpifrance qui témoigne de la solidarité de la Nation, laquelle sait accompagner ses forces vives dans les moments difficiles. Mais cette crise doit aussi nous faire prendre conscience de notre trop grande dépendance

le déficit public sera amené à se creuser largement et pourrait atteindre près de 4 % du PIB. Le groupe Les Indépendants votera, bien évidemment, ce projet de loi de finances rectificative afin de répondre à l'urgence de

s'il n'est pas question de remettre en cause les mesures proposées, que nous allons voter dans l'urgence et dans un consensus républicain, ce dernier ne doit pas nous affranchir de notre faculté de jugement et du devoir de sincérité. Surtout, la volonté de consensus ne nous interdit pas de dire aujourd'hui ce que nous disions hier. Les Français attendent de leurs élus une constance dans leurs convictions et positions. n'avons-nous cessé de dire depuis 2012 ? Qu'il fallait aller plus loin, plus vite et plus fort dans le redressement des comptes publics, sans quoi, en cas de retournement conjoncturel, notre pays ne disposerait d'aucune marge de manoeuvre budgétaire. Nous n'avons eu de cesse de le répéter, à chaque projet de loi de finances. Nous avons fait des propositions, dans la limite de ce que la LOLF et la Constitution nous permettaient. Nous n'avons jamais été entendus Le ministre de l'économie et des finances a jugé, voilà quelques jours, que la France a la chance d'avoir des finances publiques saines. Nous ne faisons pas le même constat. Personne ne le fait ! La réalité, c'est que notre pays est l'un des plus mauvais élèves de l'Union européenne. Depuis 2016, la France cumule deux distinctions : championne de l'OCDE, à la fois des prélèvements obligatoires et de la dépense publique. Si nous vous savons gré d'avoir diminué quelque peu la fiscalité des ménages et des entreprises, le Gouvernement a financé ces mesures par la dette, et donc par les impôts de demain, plutôt que par des économies. Ce n'est pas ce que nous appelons des finances publiques saines. Vous avez renoncé à toutes les économies les plus substantielles et aux réformes structurelles, les seules à même d'en dégager. La meilleure preuve étant que le déficit structurel ne diminue pas depuis des années. Les économies attendues de la réforme des retraites ont été abandonnées. En janvier dernier, le secrétaire d'État chargé des retraites avait eu le mérite de la sincérité en déclarant : « le cadrage budgétaire est clair, nous ne faisons pas ça pour faire des économies » Je rappelle que les réformes des retraites Balladur, Raffarin puis Fillon permettent d'économiser aujourd'hui 40 milliards d'euros par an. Où en serions-nous si les gouvernements d'alors n'avaient pas pris leurs responsabilités ? Ainsi, pour la première fois, une réforme des retraites constituerait une dépense et non une économie, alors même que le déficit des retraites sera de 8 à 15 milliards d'euros d'ici à 2025. Autre exemple : la suppression des 50 000 postes de fonctionnaires de l'État promise par Emmanuel Macron a été abandonnée, avec une baisse de 47 postes seulement en 2020, sur 2,6 millions de postes dans la fonction publique. Nous n'avons cessé de dire qu'Emmanuel Macron faisait la même erreur que François Hollande en repoussant sans cesse les efforts d'économies à plus tard, en fin de quinquennat. Ainsi, 19 milliards d'euros d'économies devaient succéder en 2021 et 2022 aux 14 milliards d'euros prévus en 2020. Autant dire que ces économies, déjà plus qu'hypothétiques à la veille de l'élection présidentielle, traditionnelle année des cadeaux, sont désormais improbables avec la récession qui s'annonce. Vous aviez pourtant une fenêtre de tir idéale au début du quinquennat, alors que la France bénéficiait, en 2017, d'une embellie conjoncturelle très favorable, avec une croissance économique supérieure à son niveau de 2011. Sans ces économies pour financer les baisses de fiscalité, la dette n'a cessé d'augmenter. Elle est aujourd'hui à plus de 100 % du PIB, contre 80 % en moyenne dans l'Union européenne et 61 % en Allemagne.

De même, nous sommes au vingt-quatrième rang sur vingt-sept pour le chômage, avec un taux de 8,2 % en janvier dernier contre 6,6 % dans l'Union européenne et 3,2 % en Allemagne. Seules l'Italie, l'Espagne et la Grèce font pire Enfin, s'il n'est désormais plus question du retour des comptes à l'équilibre ni même de la règle des 3 % de déficit, dans les circonstances exceptionnelles que nous connaissons, nous n'avons eu de cesse de dénoncer l'écart grandissant entre les objectifs du début et les objectifs révisés tout au long du quinquennat. Le déficit structurel n'a pas été réduit, contrairement à votre engagement initial. Avant même la crise actuelle, la promesse du retour des comptes à l'équilibre en fin de quinquennat a été progressivement abandonnée, faute d'économies. Avec un déficit de 3,1 % en 2019, la France se situe très loin de la moyenne européenne, proche des 0,5 % et donc de l'équilibre. La moitié des pays européens a des comptes excédentaires. Le déficit budgétaire français avoisine 100 milliards d'euros, tandis que l'Allemagne dégage un excédent budgétaire de 13 milliards d'euros. Pour vous, est-ce avoir des finances publiques saines ? Les pays en excédent budgétaire ont des marges de manoeuvre face à la crise actuelle, tandis que le nôtre n'en a aucune. Toutes les dépenses que nous allons engager pour sauver notre économie vont être financées par notre dette qui va s'envoler très largement au-dessus des 100 % du PIB. Nous n'avons eu de cesse, depuis 2012, de prévenir que, sans marge de manoeuvre budgétaire, la France paierait très cher le prochain retournement conjoncturel. Pour autant, madame la secrétaire d'État, monsieur le secrétaire d'État, vous pouvez compter sur nous : nous voterons ces dépenses, sans lesquelles la situation pourrait s'aggraver davantage encore, ce que nous voulons bien évidemment éviter. Si les entreprises en difficulté ne sont pas aidées, le nombre des faillites explosera et la consommation des ménages, déjà prévue en recul de 2 % en raison de la fermeture des commerces et du confinement, chutera davantage. Même si la chute de la consommation est temporaire- en de la durée des mesures de confinement -, elle pourrait devenir plus sévère à cause de la perte de pouvoir d'achat induite par la non-compensation de la perte massive des revenus. Il faut casser ce cercle vicieux au plus vite pour limiter les dégâts qui seront déjà très importants. plus que nombre de ses voisins qui ont fait les efforts nécessaires, va donc payer très cher cette crise, faute d'avoir pu assainir ses comptes. Ce quinquennat va s'achever dans la douleur, nous en sommes peinés. Au final, ce seront les Français qui le paieront, tôt ou tard. Le Président de la République a dit qu'il faudra en tirer les leçons, dont acte. Nous espérons que le Sénat sera alors davantage écouté. Encore une fois, comme pour la crise des gilets jaunes, notre seul tort est d'avoir eu raison trop tôt. Le Premier ministre nous a dit hier, ici même, non sans émotion et gravité, que l'économie allait connaître un arrêt brutal. Notre constat, c'est que la politique économique du Gouvernement n'a pas changé depuis 2012 par manque d'efforts et en raison de promesses non tenues. Pour nous, sur le plan économique, ces deux quinquennats se ressemblent, mais comment pourrait-il en être autrement ?

La séance est reprise. Par lettre en date de ce jour, le Gouvernement demande l'inscription à l'ordre du jour du samedi 21 mars, l'après-midi et, éventuellement, le soir, sous réserve de leur dépôt, des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances rectificative pour 2020 et des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ou l'examen en nouvelle lecture de ces projets de loi. Nous lui donnons acte de cette demande. Je propose que la durée de la discussion générale sur ces deux textes soit fixée à quarante-cinq Il n'y a pas d'opposition ? ... En cas de nouvelle lecture, mes chers collègues, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance serait fixé à l'ouverture de la discussion générale. pas d'observation ? ... Il en est ainsi décidé. Nous passons à la discussion des articles du projet de loi de finances rectificative pour 2020.

immédiatement rendu disponible ce volant de 5 000 euros qui permettra, dans les semaines qui viennent, de défiscaliser une partie des heures supplémentaires. Je peux vous

... que la fameuse prime pour les « gilets jaunes » représentait à peu près 400 euros. Le dispositif que nous proposons est beaucoup plus massif, pour encourager celles et ceux qui sont aujourd'hui en première ligne, et davantage incitatif pour les entreprises. Le Medef l'a d'ailleurs

d'un texte récent, la loi Pacte, pour rendre l'intéressement obligatoire dans toutes les entreprises de plus de dix salariés. Je suis donc très favorable aux principes de répartition, d'encouragement et de récompense qui sous-tendent l'intéressement et la participation.

monsieur le ministre,

Je pense même que cette mesure, et ma collègue Agnès Pannier-Runacher l'a dit précédemment, est utile pour accompagner un plan de relance, et nous sommes évidemment ouverts à l'idée de travailler ensemble dans ce cadre, notamment- mais pas seulement -pour avancer et faire en sorte que, dès que notre économie repartira, nous puissions l'accompagner de la façon la plus forte possible.

Nous les assortissons de 300 milliards d'euros de garanties, ce qui est massif, même si nous avons tous l'espoir que ces garanties apportées à des prêts aux entreprises ne donneront pas lieu à couverture, ce qui serait la meilleure des nouvelles pour notre économie.

sanitaire. Dans ce cadre, nous pourrions, et c'est la raison pour laquelle j'appuie la demande de retrait de ma collègue Agnès Pannier-Runacher, nous retrouver utilement dans les prochains jours ou les prochaines semaines pour travailler sur ce dispositif et éventuellement sur d'autres pistes. Nous aurons

devait y avoir un dépassement du plafond des 5 000 euros, tel qu'il est prévu par les dispositions actuellement en vigueur, nous connaissons, vous et moi, la capacité du Parlement, surtout dans ces conditions, à prendre des mesures rétroactives. J'appuie donc la demande de retrait

Mon collègue du CNRS Bruno Canard, directeur de recherche, travaille depuis très longtemps sur la famille de virus à laquelle appartient celui

l'hiver prochain, parce qu'on peut redouter que ce virus soit, comme celui de la grippe, saisonnier. Nous devons travailler dès maintenant, et en toute urgence, sur les voies médicamenteuses pour guérir ce virus,

le montant ici proposé- 50 millions d'euros -semble raisonnable au regard de la budgétisation traditionnelle du crédit d'impôt recherche qui doit être, si je ne m'abuse,

l'avis du Gouvernement ?

conséquent, des masques sont produits dans le monde, des pays s'en procurent et, en France, les collectivités souhaitent aider le Gouvernement à relever le défi. Aidez-nous

; en effet, nous considérons que des acheteurs qui ont eu la capacité de bloquer des contingents de masques ont fait un effort et, compte tenu de l'usage de ces masques, nous ne bloquerons pas ces importations.

mais, pour ceux qui ont juste un emploi et un petit salaire, c'est déjà fait ! Tous ceux qui sont mis au chômage partiel, avec 84 % de leur salaire, commencent à payer !

hier, une séance, au cours de laquelle la ministre Pénicaud a complètement remis en cause ce qui restait du code du travail, au désavantage des salariés ; ça, on peut le faire très vite, il n'y a aucun problème

ils ne sont pas en télétravail. L'amendement présenté par notre collègue Savoldelli vise un revenu fiscal de référence supérieur à 250 000 euros par an et on ne propose pas une spoliation, il s'agit de passer de 3 %

votons, avançons. Montrons que le Sénat sait être à la hauteur de ses responsabilités et sait aussi trancher vite les débats. Il y a une urgence sanitaire, ces mesures sont attendues ; votons et avançons. Je

mais ayons-le quand même ! Ne croyons pas que nos concitoyens ne débattent pas, même quand ils sont confinés.

Je ne vois pas de lien immédiat entre cet amendement et l'action que nous menons contre le coronavirus. Chaque article de ce projet de loi a vocation

A annexé. Avant de mettre aux voix l'ensemble de la première partie du projet de loi de finances rectificative pour 2020, je rappelle que, en application de l'article 42 de la loi organique

les entreprises et les indépendants qui auraient rencontré des difficultés fortes entre le mois de mars 2019 et le mois de mars 2020, notamment pour les entreprises réalisant un chiffre d'affaires de moins de 1 million d'euros.

Chacun sait ici que, dans la crise que nous traversons, l'une des situations les plus dramatiques est celle des personnes les plus précaires, en particulier les sans-abri. Je le constate notamment en tant qu'élu parisien : aujourd'hui, l'une des principales tâches de la Ville de Paris est de mobiliser l'ensemble des acteurs pour venir en soutien aux sans-abri qui errent dans les rues. Ils voient certaines structures fermer et des lieux de distribution alimentaire diminuer leurs prestations ; enfin, ils se trouvent souvent en grande difficulté et peuvent, de ce fait, être d'autant plus victimes de l'épidémie. Les responsables du Secours populaire nous disaient aujourd'hui qu'il leur faudrait en urgence 10 millions d'euros pour faire face aux besoins immédiats, d'autant plus que les dons sont rendus plus difficiles actuellement.

d'euros. Nous savons que l'ensemble des lieux de culture ont dû fermer leurs portes et que leur équilibre économique est à l'évidence très gravement mis en péril.

librairies, notamment aux librairies indépendantes. Nous savons que leur équilibre économique est fragile, que leurs marges sont très réduites, que la crise sanitaire

n'ouvrent pas seulement leurs rayons alimentaires, mais aussi leurs rayons de librairie, ce qui crée à l'évidence une concurrence tout à fait déloyale. C'est pourquoi nous proposons un fonds de soutien aux librairies de France : nous savons que c'est un enjeu

monsieur le ministre,

utile, dans le cadre des plans de continuité d'activité, à ce qu'un certain nombre de fonctions soient préservées : je pense notamment aux fonctions de paye, notamment des agents publics, mais aussi des allocations et des minima sociaux. En effet, il serait absolument dramatique qu'un ralentissement de l'activité de nos services se traduise par l'impossibilité de verser telle ou telle allocation.

à cette urgence. Je ferai deux remarques pour finir. Tout d'abord, je réitère la demande de retrait en soulignant bien qu'il n'y a pas là d'appréciation sur le fond. Nous partageons le le constat qu'une aide sera très probablement nécessaire dans les temps qui viennent pour ce secteur, mais nous voulons l'élargir et la maintenir dans les dispositifs du plan de relance. Ma seconde remarque concerne les collectivités territoriales.

disposent- c'est un chiffre global qui, comme tous les chiffres globaux, ne vaut que pour sa globalité, et non pas collectivité par collectivité -d'une trésorerie de 44 milliards d'euros. Il y aura certainement des impacts sur les collectivités locales, mais nous pourrons les traiter dans un texte qui ne relève pas de la même urgence

Le sujet mérite que l'on s'y arrête un instant. Je pense notamment à l'amendement sur le fonds de soutien aux librairies. C'est typiquement l'exemple d'un secteur qui subit, si je puis dire, la double peine : il y a d'abord l'absence de chiffre d'affaires, mais, en plus, la concurrence

des points de livraison et poursuivre leur activité en e-commerce. On a élaboré dimanche dernier un guide de bonnes pratiques sur la livraison des repas à domicile. Cela peut paraître paradoxal, mais on va avoir besoin de cuisines qui tournent pour aller livrer

à un communiqué de presse commun explicitant comment on peut reprendre le travail. Il ne s'agit évidemment pas d'exposer les personnels de chantier. Cela doit se faire de manière raisonnée, probablement en diminuant la voilure, mais, en tout état de cause, on a aussi besoin de l'intervention de ces experts dans différentes situations. C'est ce sur quoi nous travaillons. Il y a effectivement

inquiets. La question est toujours la même : comment vivre au jour le jour ? Il faut trouver des mesures, peut-être avec Pôle emploi Spectacle, peut-être en revoyant les règles qui s'appliquent à l'intermittence, car un grand nombre de structures sont profondément menacées. C'est la réalité ! C'est immédiat ! Si on ne vote pas ces amendements, il faut de toute façon trouver des solutions. J'en profite pour parler aussi de la question des librairies. J'entends bien ce que vous dites, monsieur le rapporteur général.

est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote. Je partage bien évidemment les observations de M. le rapporteur général sur ces amendements, mais je voulais revenir quand même sur le premier, qui concerne l'aide alimentaire,

qui ont vocation à payer 85 % de la dépense engagée par l'État. Malheureusement, notre organisation et notre administration ont été défaillantes et incapables de répondre au cahier des charges que nous nous étions fixé à nous-mêmes pour obtenir ces remboursements. C'est un problème central. Aujourd'hui, l'aide alimentaire va être en difficulté pour plusieurs raisons. D'abord, certains présidents d'association ont organisé un retrait des bénévoles, qui font partie des populations les plus âgées de notre pays, et qui, légitimement, peuvent s'inquiéter du contact avec le public.

sera attentif à cette question, qu'il a les moyens d'y répondre immédiatement, quitte à nous demander ensuite de régulariser les mesures budgétairement. En tout cas, 5,5 millions de personnes dépendantes aujourd'hui de cette aide alimentaire

Je reviens sur le dossier des petites librairies, sans répéter les arguments qui ont été exposés ici, auxquels je m'associe absolument. Plusieurs libraires m'ont contacté en me disant qu'ils avaient des stocks

absolument immense. Vous le savez bien, Amazon finance les frais d'envoi- quand vous achetez, c'est gratuit -, grâce à ses marges arrière, en intégrant le coût des expéditions dans ces marges. Les petits libraires, bien évidemment, ne peuvent pas recourir à cette pratique. Une mesure de justice serait soit d'offrir une baisse

(DMTO) risquent d'être moins importants cette année et, en tout cas, de reculer dans le temps. Il faut donc aussi prendre en compte cette dimension financière, qui me paraît tout à fait importante. Ensuite, nous avons beaucoup parlé de la question des librairies. C'est vrai que nous cherchons tous des moyens pour que, dans cette période qui permet à beaucoup de Français de lire, les librairies puissent en profiter autrement qu'en ouvrant leur magasin,

Ce dispositif, tel qu'il est prévu, en permettant à un certain nombre de structures de commercialiser des biens qui ne sont pas des biens de première nécessité, parce qu'ils ont les moyens de le faire- je ne parle pas uniquement des plateformes, car il y a aussi la grande distribution

sanitaire. Les 5 millions de bénéficiaires de l'aide alimentaire font partie de ceux que l'on appelle les personnes vulnérables. Si on laisse les associations dans la situation dans laquelle elles sont,

Merci ! Je crois que ce débat n'était pas inutile pour des perspectives futures. La parole est sont, vous l'avez dit vous-même, des amendements d'appel, mais d'appel d'attention. Nous avons évoqué les uns et les autres d'autres sujets qui méritaient cette même attention. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Je peux vous garantir de nouveau que l'ensemble des moyens que nous pouvons mobiliser le sont pour accompagner tous les secteurs. Vous avez cité des secteurs qui rencontrent des difficultés particulières, il faut le souligner, mais il y en a d'autres. Nous veillerons évidemment à ce que les plus fragiles soient aussi

Nous avons aussi mis en avant, et nous venons de le faire, un certain nombre de manques, car ce projet de loi est lacunaire. Il en appelle d'autres. Nous avons souhaité créer des fonds de soutien, et chacun a pu exprimer sa solidarité à l'égard de secteurs particulièrement fragiles : la culture, les librairies, l'aide alimentaire.

veux m'expliquer sur les annonces que nous avons faites en matière de financement des hôpitaux. Le Président de la République s'est engagé sur un premier déblocage de fonds de 2 milliards d'euros. Nous verrons si nous devons abonder ces fonds en fonction de l'évolution de la situation, bien évidemment.

: nous n'avons pas besoin, d'un point de vue totalement matériel et en droit, de vous présenter maintenant une loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour pouvoir ajouter des crédits. Je le dis en apportant une précision

L'Ondam est un objectif. Il n'est pas une norme de dépenses en soi, et il n'a pas le caractère impératif que peuvent avoir certains crédits, certains programmes du budget de l'État. Ce sont bien 2 milliards d'euros nouveaux

Ce sont là les réponses aux premières demandes qui nous sont remontées. J'imagine qu'il y en aura d'autres. Pour anticiper sur une éventuelle question, je précise qu'il s'agit essentiellement d'investissements, en tout cas d'achats de matériel,

pour explication de vote. J'informe notre collègue Fabien Gay que le préfet de Seine-Saint-Denis vient, comme il le fait chaque fois, de réquisitionner des gymnases dans les collectivités locales. J'ai envie de dire que c'est mieux que rien.

à accepter toutes les mesures budgétaires exceptionnelles quitte à oublier les impératifs du traité budgétaire en vigueur. Et même la Banque centrale européenne n'exclut plus le rachat des dettes publiques des États.

vote. « Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. » Ce n'est pas Karl Marx qui a dit cela ; c'est le président Macron

que vous veniez sur nos positions. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui est pourtant un fervent adepte des privatisations, vient d'annoncer qu'il était d'accord pour des nationalisations totales ou partielles de certains pans de notre économie. J'ai entendu avec plaisir notre

tandis que les taux Eonia et Euribor sont singulièrement bas, voire négatifs, faisant en sorte que les taux d'intérêt ne sauraient être aussi élevés qu'ils peuvent l'être aujourd'hui.

pour accompagner les entreprises qui seraient confrontées à des difficultés, et Bpifrance garantit 90 % des prêts bancaires, ce qui donne un confort sur le risque très élevé limite l'évolution des taux.

donc bien falloir changer la manière dont on utilise ces énormes mannes financières. Il va bien falloir repenser la manière dont on contrôle les taux de crédit, à qui on les donne, pour faire quoi, sur quels critères, etc. C'est comme pour le chômage partiel.

rédigé, l'article 4 du projet de loi prévoit que la garantie ne peut être accordée à des prêts bénéficiant à des entreprises faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire. Or, à la différence des entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire, celles qui font l'objet d'une procédure de sauvegarde ne sont pas en cessation de paiements. de paiements. Cette procédure « est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ». Exclure ces entreprises du bénéfice de la garantie de l'État serait donc contre-productif : alors même qu'elles présentent non pas des problèmes de liquidité, mais uniquement des difficultés temporaires, elles seraient fortement pénalisées. Il est donc Il est donc impératif de prévoir que les entreprises en sauvegarde puissent bénéficier de ce dispositif. Dans le cas contraire, le nombre de faillites augmenterait fortement, à rebours des engagements du Président de la République.

12 est retiré.

pleinement son contrôle sur ces engagements de l'État. Ce raisonnement vaut aussi bien pour le fonds de solidarité que pour le mécanisme de garantie des prêts. prêts. Il est vrai que l'Assemblée nationale, sur proposition du président de sa commission des finances, a prévu un comité de suivi. Ce comité est sans doute utile, mais les circonstances

de l'évolution de la situation économique cette année. Enfin, comme je l'ai indiqué à M. Féraud, même s'il ne s'agit là que d'un chiffre global, nous savons que les collectivités territoriales dans leur ensemble disposent aujourd'hui d'une trésorerie de 44 milliards d'euros. Par ailleurs, d'autres éléments de leurs recettes, comme les dotations, sont garantis par la loi de finances pour 2020, contrairement aux entreprises qui voient leur chiffre d'affaires, donc leurs recettes, s'écrouler cette année. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'impact et je ne sous-estime pas le fait

position. D'aucuns ici pourraient s'arroger l'esprit de responsabilité au détriment d'autres sensibilités politiques. C'est vrai ! Nous ne le faisons pas et nous avons raison,

qui sont devant nous et des désaccords normaux dans le débat démocratique. Il s'agissait aujourd'hui de tenter de parer à des situations d'urgence : urgence sociale, urgence sanitaire, urgence aussi

un chèque en blanc : l'impact financier de la crise actuelle sera considérable, on ne sait pas le mesurer aujourd'hui et de nombreux points devront être traités demain. Le ministre de l'action et

de la concurrence dans certains secteurs de la distribution, mais je pense que d'autres reviendront sur le sujet. En tout cas, ce train de mesures me paraît positif et aujourd'hui adapté, mais il méritera sûrement d'être amélioré, amendé et renforcé dans les semaines et les mois à venir.

La crise sanitaire conduit à un choc de demande, en raison des contraintes de déplacement, des restrictions d'ouverture des commerces et des capacités de travail des entreprises et à un choc d'offre du fait des défaillances multiples des chaînes d'approvisionnement à court terme, l'impact sur les finances publiques sera particulièrement lourd, avec une baisse des recettes due à la contraction de l'économie, d'une part, et une augmentation des dépenses due aux mesures de soutien exceptionnel, d'autre part. que nous venons d'examiner vise à acter cette dégradation brutale des finances publiques. Il permet au Gouvernement de débloquer les fonds nécessaires au financement des mesures qui seront rapidement déployées, notamment concernant le chômage partiel et la garantie apportée par l'État pour les crédits alloués aux entreprises en difficulté.

de la demande française comme étrangère, qui ne sont pas acquis, si bien que la dégradation du cadre macroéconomique pourrait être plus marquée que prévu actuellement. Cette dernière hypothèse devra sans doute être réexaminée dans les semaines qui viennent.

Le deuxième enseignement tient au fait que nombre d'entre vous ont exprimé la conviction, que nous pouvons partager au vu de la situation, que ces mesures en appelleront peut-être d'autres et qu'un certain nombre de questions n'ont pu trouver de réponses suffisamment précises aujourd'hui,

et, éventuellement, après-midi, de l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ou de l'examen en nouvelle lecture de ce texte, qui avaient été initialement inscrits le samedi 21 mars.

Acte est donné de cette demande. Mes chers collègues, comme nous en avions décidé le principe lors de notre dernière conférence des présidents, il est essentiel que, dans les circonstances particulières où nous nous trouvons placés, la mission de contrôle du Sénat puisse continuer de du Sénat puisse continuer de s'exercer. C'est pourquoi je vous propose de maintenir le principe d'une séance de questions d'actualité le mercredi à selon des modalités particulières d'organisation qui vous seront rapidement communiquées. Les présidents de groupe ont été consultés et ont donné leur accord de principe ; les modalités pratiques seront définies en lien avec eux. Ainsi, notre prochaine séance de questions d'actualité aura lieu mercredi 25 mars à quinze heures. Y a-t-il des observations ?